Monsieur le président,

La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 22 mai 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. Mes chers collègues, par lettre en date du mercredi 22 mai, M. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains, a demandé le retrait de la proposition de loi portant adaptations législatives aux spécificités des territoires d'outre-mer soumis à une pression migratoire importante, inscrite à l'ordre du jour du mercredi 12 et du jeudi 13 juin 2019. Acte est donné de cette demande. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la conservation

Monsieur le président, madame la présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, chère Catherine Morin-Desailly, monsieur le président de la commission des finances, cher Vincent Éblé,

monsieur le rapporteur pour avis de la commission des finances, cher Albéric de Montgolfier, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous nous rappelons tous où nous étions, le lundi 15 avril au soir, quand nous avons vu pour la première fois les images de Notre-Dame embrasée. C'était il y a exactement six semaines. Plus qu'un monument, plus qu'une cathédrale, elle est une part de la France, de son histoire, de son identité. Elle est une part de nous-mêmes. Voilà qui explique que ce feu nous ait touchés au coeur. Voilà qui explique que nous ayons tressailli en imaginant le pire, en imaginant que nous assistions, peut-être, aux derniers instants de Notre-Dame de Paris. Voilà qui explique, aussi, l'extraordinaire mobilisation qui a suivi, si tant est qu'on puisse expliquer une mobilisation d'une telle ampleur. Ce fut, d'abord, la mobilisation de femmes et d'hommes qui, parfois au péril de leur vie, ont arrêté l'embrasement et sauvé les oeuvres exceptionnelles présentes dans la cathédrale : les sapeurs-pompiers de Paris, aidés et renforcés par leurs collègues des autres départements d'Île-de-France, mais aussi les policiers, les agents du ministère de la culture, de la Ville de Paris et du diocèse. Je veux très sincèrement, une nouvelle fois, les remercier pour leur engagement. Si les voûtes restent encore très fragilisées, l'édifice est aujourd'hui largement sauvé. Nous le devons à leur professionnalisme, à leur dévouement, à leur courage. Cette mobilisation, c'est aussi celle d'experts, d'institutions et d'entreprises dont les promesses de dons et les propositions d'aide en compétences se sont multipliées. Surtout, c'est une mobilisation populaire. Des centaines de milliers de dons de particuliers ont afflué de toutes parts, de France et de par le monde. Aujourd'hui encore, ils continuent de nous parvenir. Il fallait créer un cadre pour les accueillir, pour accompagner, encourager, encadrer cet élan de générosité, pour assortir cette ferveur exceptionnelle d'un dispositif exceptionnel. C'est le sens du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. Oui, nous restaurerons Notre-Dame de Paris ! Le Président de la République a fixé un objectif : cinq ans. C'est un délai ambitieux et volontariste, qui permet de motiver les équipes et de mobiliser l'ensemble des acteurs concernés. Pour autant, dans cette tâche qui nous attend, nous ne confondrons jamais vitesse et précipitation. Nous devons offrir à Notre-Dame une restauration à la hauteur de sa splendeur, à la hauteur de ce qu'elle symbolise. Sur un certain nombre de points, il y a urgence à intervenir ; sur d'autres, nous devrons prendre le temps de la réflexion.

Ce sont les dons pour Notre-Dame qui ont abondé vite ! Et il fallait pouvoir y répondre tout aussi vite. C'est ce que nous avons fait, et je l'assume pleinement. Que nous aurait-on dit si nous avions laissé fleurir les arnaques, les faux sites internet, les fausses cagnottes en ligne, si nous n'avions pas lancé la souscription nationale, alors que Notre-Dame appartient à la Nation tout entière ? Que nous aurait-on dit si nous n'avions rien fait ? On nous aurait dit que l'État manquait à sa mission, et on aurait eu raison de nous le dire, car c'est à l'État d'intervenir pour protéger ce patrimoine commun. Ce n'est pas un péché d'orgueil et ce n'est pas déplacé. C'est la responsabilité de l'État, à la fois, d'encadrer la souscription nationale dédiée, en fixant, par la loi, les règles qui lui sont applicables, et d'apporter des garanties de sécurité et de transparence aux centaines de milliers de donateurs français ou étrangers. Cette transparence, nous la leur devons. Je veux les remercier, très sincèrement, pour leur générosité. Ils ne seront pas trahis : leurs dons iront à Notre-Dame de Paris, uniquement et intégralement, à sa conservation, à sa restauration et à son entretien, à court et moyen terme. Nous y veillerons ; soyez-en assurés. Certains avancent l'idée que nous aurions déjà collecté trop de fonds, plus qu'il n'en faut pour restaurer la cathédrale. Mais si certains dons nous sont déjà parvenus, d'autres sont encore en attente de concrétisation. En outre, le coût total des travaux n'a pas encore été chiffré. En effet, pour l'instant, les travaux portent seulement sur la mise en sécurité de l'édifice, qui reste, je veux le redire, fragile au niveau de la voûte. à cette occasion de remercier très sincèrement, pour leur dévouement et leur réactivité, les entreprises, qui, dès le lundi soir, avec les services du ministère de la culture, ont entrepris un travail exceptionnel pour sauvegarder l'essentiel. Merci à elles et à toutes leurs équipes,

Ce n'est qu'ensuite que nous passerons à la phase de diagnostic, puis à la restauration elle-même. Dans ces conditions, il est prématuré d'affirmer que nous aurions des surplus à gérer. Pour opérer cette souscription nationale, outre les versements directs à l'État, nous pouvons compter, depuis le 16 avril, sur la mobilisation de trois fondations reconnues d'utilité publique- la Fondation de France, la Fondation du Patrimoine la Fondation Notre-Dame -et du Centre des monuments nationaux, opérateur du ministère de la culture. Je veux les en remercier.

Dans un même souci de transparence quant à l'emploi des fonds collectés, un comité de contrôle sera mis en place. Il réunira le Premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions chargées des finances et de la culture du Sénat et de l'Assemblée nationale.

ni les droits du culte affectataire, c'est-à-dire la répartition des prérogatives et des responsabilités entre l'État et l'Église catholique. L'intégralité des dons passera ainsi par la souscription nationale, à l'exception de ceux qui ont spécifiquement pour objet de financer la restauration des biens appartenant au diocèse ou, plus généralement, les besoins relevant de l'exercice du culte. Cette loi, je le disais, doit garantir la transparence de la souscription nationale ; elle doit aussi en fixer les règles. En ce qui concerne les particuliers, la loi introduit un dispositif fiscal spécifique pour accompagner leurs dons. Je tiens à saluer le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, ainsi que le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, pour le travail que nous avons réalisé en étroite collaboration. Dans la limite de 1 000 euros, le projet de loi porte de 66 % à 75 % le taux de réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons et versements effectués par les particuliers en faveur du Trésor public, du Centre des monuments nationaux et des trois fondations que j'ai mentionnées. Ce dispositif, je le rappelle, ne concerne que les particuliers et les entreprises unipersonnelles. Il a été conçu de manière à couvrir les dons du plus large nombre de Français. Il est précisément limité, dans le temps, puisque cet avantage fiscal ne concerne que les dons effectués entre le 16 avril et le 31 décembre 2019, et dans les montants, puisque le plafond de don éligible à la réduction fiscale est fixé à 1 000 euros. Ces limites n'empêchent de donner ni au-delà de cette date ni au-dessus de ce plafond. Seulement, dans ce cas, l'avantage fiscal associé au don sera celui de droit commun. Les collectivités territoriales et leurs groupements pourront aussi participer au financement des travaux, au-delà de leur périmètre de compétence territoriale. L'article 4 lève toute incertitude éventuelle tenant aux règles habituelles de compétence ou à la condition d'intérêt local. Le ministre de l'action et des comptes publics aura l'occasion de le redire : les dépenses des collectivités en faveur de Notre-Dame seront considérées comme des dépenses d'équipement. Elles ne seront donc pas prises en compte pour appréhender le plafond annuel d'évolution des dépenses de fonctionnement de 1,2 %. Sur tous ces sujets, je le disais, nous irons vite, mais nous ne nous précipiterons pas. La restauration ne se fera pas dans la hâte. Elle doit être à la hauteur, je l'ai dit et je le répète, de la splendeur de Notre-Dame de Paris. Nous devons faire en sorte que cette restauration soit exemplaire. Nous saurons prendre en compte l'avis des professionnels du patrimoine, des conservateurs, des architectes, des historiens, des universitaires et de tous ceux qui oeuvrent à l'entretien, à la conservation et à la restauration de nos monuments. Nous saurons les écouter et nous saurons leur faire confiance.

Nous sommes en train de réfléchir à l'organisation optimale pour mener à bien ce chantier au regard des objectifs fixés. Le choix d'organisation n'est pas encore finalisé, mais notre réflexion avance. Nous nous donnons notamment la possibilité de créer un établissement public nouveau à cet effet. Quel que soit le choix d'organisation retenu, il permettra de prendre en compte l'avis des professionnels du patrimoine au travers d'un conseil scientifique, qui sera le garant de la qualité scientifique et historique de la restauration. Quoi qu'il en soit, je veux affirmer devant vous trois points capitaux. Premièrement, la maîtrise d'oeuvre de ce chantier sera effectuée, dans les règles de l'art, par les architectes en chef des monuments historiques, en l'occurrence Philippe Villeneuve, qui a la charge de Notre-Dame de Paris. comme il se doit dans un chantier de cette ampleur, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sera régulièrement consultée sur l'avancée des travaux et les choix de restauration.

quel que soit le choix d'organisation qui sera retenu, il devra permettre de prendre en compte les intérêts légitimes des principales parties prenantes intéressées à la restauration, notamment le diocèse et la Ville de Paris. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, si aucune opération de restauration de monument historique n'avait encore donné lieu à une telle adaptation législative, c'est parce que nous sommes face à une situation exceptionnelle. Le chantier qui s'annonce est ambitieux et unique. Pour le mener au mieux, nous voulons nous donner la possibilité d'assouplir certaines dispositions, essentiellement de procédure, mais il va de soi que les assouplissements aux législations en vigueur seront strictement proportionnés aux besoins du chantier. Il n'est pas question de se servir de la restauration de Notre-Dame pour piétiner le droit français et européen du patrimoine, de l'environnement, ou de l'urbanisme. Cela n'a bien évidemment jamais été l'intention du Gouvernement. Je veux le dire et le redire : en tant que ministre de la culture, je serai inlassablement le garant de la protection du patrimoine et j'aurai à coeur de mobiliser l'ensemble des ministres concernés. Le travail interministériel des prochaines semaines nous permettra de définir, ensemble, les assouplissements et les adaptations à prévoir, qui porteront essentiellement sur des questions de procédure, sans remettre en cause le fond des législations applicables. À chaque instant, nous imposerons la préservation de l'intérêt historique, artistique, architectural et symbolique du monument. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, fallait-il une loi pour engager la restauration de Notre-Dame ? Voilà sans doute l'une des questions que nous nous sommes tous posées lorsque, seulement neuf jours après avoir été saisis d'effroi devant les ravages qu'un funeste incendie causait à la cathédrale, ce texte a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Sans doute faut-il préalablement répondre à plusieurs autres questions pour pouvoir répondre correctement à celle-ci. Premièrement, fallait-il faire appel à la générosité du public pour financer les travaux de restauration de Notre-Dame, monument historique à la charge de l'État ? La mission d'information sur le mécénat culturel, qu'a présidée notre collègue Maryvonne Blondin et dont j'ai été le rapporteur, avait alerté l'an passé sur les effets d'éviction que pouvait entraîner le recours de l'État à des procédures de souscription pour la restauration des monuments historiques qui lui appartiennent. Certes, la situation m'apparaît un peu différente dans le cas présent, mais convenons que l'élan de générosité du public a précédé l'annonce de la souscription nationale. Je note que le ministre de la culture s'est par ailleurs engagé à ce que l'État prenne en charge le surcoût si le produit de la souscription se révélait insuffisant pour couvrir le coût des travaux. Il a indiqué que l'État était prêt à assurer le financement au-delà des crédits inscrits sur le programme 175 et a garanti que sa participation ne se ferait pas au détriment d'autres chantiers et d'autres monuments. Ce sont des engagements importants, qu'il nous appartiendra évidemment d'évaluer dans les années à venir. Deuxièmement, cette souscription nationale devait-elle être lancée par le biais d'une loi ? Il est clair qu'un décret aurait été tout à fait suffisant d'un point de vue juridique. Reconnaissons néanmoins que ce choix donne l'occasion d'un débat public au sein de la représentation nationale sur le sujet de la restauration de Notre-Dame, ce qui est tout à fait souhaitable au regard de l'enjeu soulevé par la perspective de cette restauration et les polémiques qu'elle suscite. Troisièmement, la majoration du taux de la réduction d'impôt accordée aux particuliers pour les dons qu'ils effectuent au titre de la souscription nationale est-elle vraiment utile ? Les dons et promesses de dons ont afflué avant même l'annonce de cette majoration, ce qui laisse à penser que l'incidence de celle-ci sur l'acte de don est négligeable. C'est avant tout l'émotion créée par un tel événement qui motive les donateurs. C'est d'ailleurs ce que semble indiquer le ralentissement des dons versés aux fondations reconnues d'utilité publique. Pour avoir été le rapporteur, l'an passé, de la mission d'information sur le mécénat culturel, j'ai pu constater combien nous disposions déjà d'un dispositif fiscal particulièrement attractif, que beaucoup d'autres pays nous envient, au point de s'en être largement inspirés pour élaborer leur propre législation en matière de soutien au mécénat. Limitée aux dons des particuliers à hauteur de 1 000 euros, cette majoration exceptionnelle du taux de 9 points est avant tout symbolique. C'est un moyen de remercier nos compatriotes pour leur générosité et de reconnaître le caractère exceptionnel du chantier de Notre-Dame. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Sans doute nous faudra-t-il même garder ce cas à l'esprit dans quelques mois, lorsque des propositions de remise en cause de notre régime de mécénat pourraient venir sur la table à l'occasion du prochain projet de loi de finances. Quatrièmement, le recours aux ordonnances ne trahit-il pas les incertitudes et la précipitation du Gouvernement, alors que celles-ci portent sur des sujets qui auraient justifié que le Gouvernement prenne davantage son temps ? Sur les neuf articles du projet de loi, deux articles habilitent le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances. Alors que le Parlement regarde toujours avec beaucoup de méfiance les articles d'habilitation, qui réduisent significativement sa capacité à procéder à un examen attentif des dispositions qui lui sont soumises, les deux articles d'habilitation du présent texte portent sur des sujets à la fois majeurs et fort peu consensuels la création d'un établissement public spécifiquement chargé de la restauration de Notre-Dame, d'une part, et l'octroi de dérogations aux législations existantes pour faciliter la réalisation de ce chantier, aussi exceptionnel soit-il, d'autre part. Sans compter que ces deux dispositions ont été interprétées par beaucoup comme des marques de défiance à l'égard, à la fois, des capacités propres au ministère de la culture à conduire lui-même ce projet, compte tenu du souhait qui transparaît de nommer Jean-Louis Georgelin à la tête du futur établissement public,

mais aussi le Centre des monuments nationaux et l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture. Alors qu'une circulaire du Premier ministre devait prochainement être publiée, demandant qu'aucun établissement public ne soit créé sans qu'un autre soit préalablement supprimé, on peine à comprendre la volonté de créer un nouvel établissement. Au demeurant, il faut reconnaître que cette solution a été utilisée à de multiples reprises par le passé, avec succès : le Grand Louvre, la bibliothèque François-Mitterrand, ou encore le musée du Quai Branly Elle peut constituer une garantie de transparence pour un chantier exceptionnel et financé d'une manière particulière, en l'occurrence une souscription. Elle peut donc être acceptable, sous réserve d'en encadrer les missions et le fonctionnement. C'est ce que nous avons cherché à faire en commission, en précisant le caractère administratif de l'établissement, en le plaçant sous la tutelle du ministère de la culture et en rappelant que la maîtrise d'oeuvre serait conduite sous l'autorité des architectes en chef des monuments historiques. Ce qui n'est pas acceptable, en revanche, c'est de laisser ainsi planer l'ambiguïté sur la solution qui sera retenue par l'État, entre les moyens qu'il a déjà à sa disposition et la création d'un nouvel établissement public. C'est se défier du Parlement et faire fi de la nécessaire intelligibilité de la loi ! Très bien ! De la même manière, les dérogations aux règles de droit commun prévues à l'article 9 nous semblent inutiles si l'objectif est de gagner du temps sur les démarches administratives. effet, les demandes d'autorisation concernant Notre-Dame pourront parfaitement être traitées de manière prioritaire par les services de l'État moyennant des instructions en ce sens. Il est absurde de se laisser enfermer dans le délai de cinq ans annoncé par le Président de la République s'il doit conduire à rogner sur la qualité du chantier, dont nous savons tous qu'il sera observé par le monde entier, ou à écarter nos entreprises et nos compagnons spécialisés dans la restauration du patrimoine, que nous souhaitons mettre en valeur à l'occasion de ce chantier exceptionnel. Aucune cathédrale n'est restaurée pour seulement une dizaine d'années ! Il faut se donner le temps de la réflexion et consulter le plus largement possible les experts. Le délai de cinq ans ne doit pas être autre chose qu'une ambition au service d'une mobilisation. Nous pensons également que ces dérogations pourraient se révéler dangereuses si l'objectif est de permettre à l'État de s'affranchir de règles que les autres propriétaires doivent mettre en oeuvre lorsqu'ils conduisent des projets de restauration, quand bien même leur ampleur est différente.

Nous estimons, dans ces conditions, que le risque de jeter le discrédit sur l'ensemble de notre législation est énorme et constituerait, à coup sûr, un précédent désastreux- je pèse mes mots -pour l'avenir. Tout à fait ! C'est pour cette raison que nous avons supprimé l'article 9 lors de l'examen du projet de loi en commission, la semaine dernière. Oui, le chantier de Notre-Dame est un chantier exceptionnel. Oui, le chantier de Notre-Dame est un chantier emblématique. C'est la raison pour laquelle il doit être un chantier exemplaire. N'oublions pas que la présence de Notre-Dame a constitué un élément déterminant dans l'inscription du bien « Paris, rives de la Seine » sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, ce qui implique un certain nombre d'obligations pour notre pays dans la manière dont nous le restaurons. Nous n'avons pas besoin d'un geste architectural pour que Notre-Dame devienne « plus belle encore ». Notre-Dame a toujours été un joyau. Elle a une histoire, dont nous ne saurions faire abstraction ; qu'on le veuille ou non, Viollet-le-Duc en fait partie. Par chance, les relevés de la charpente et de la flèche existent, les statues et le coq qui ornaient la flèche ont été sauvés. pourquoi écarter d'office l'option d'une restauration fidèle, alors même que c'est probablement celle qui permettrait de gagner le plus de temps ? C'est vrai ! Avons-nous vraiment besoin de laisser notre marque sur la cathédrale ? Si marque il doit y avoir, doit-elle vraiment porter sur la flèche ? Il me paraît primordial que les décisions qui seront prises soient parfaitement documentées pour permettre aux générations futures de comprendre ce qui nous a amenés à ces solutions. Nous devons aussi mettre à profit ce drame autant que faire se peut. S'il doit bien y avoir un « avant » et un « après » le 15 avril, selon vos mots, monsieur le ministre, cela concerne moins l'esthétique d'une nouvelle flèche que la manière dont nous percevons notre patrimoine et dont nous le protégeons. Le chantier de Notre-Dame doit devenir une vitrine de notre régime de protection patrimoniale, une vitrine de nos savoir-faire dans ce domaine, bref une vitrine à la hauteur de notre réputation Dans un article paru la semaine dernière, le Sénat était décrit comme « le dernier rempart de la démocratie patrimoniale en danger ». Nous aurons à coeur de défendre cette position au cours de l'examen de ce projet de loi. De ce point de vue, les amendements que le Gouvernement a déposés, qui tendent purement et simplement à rétablir le texte de l'Assemblée nationale sans prendre en compte un seul des

exceptionnelle de la réduction d'impôt sur le revenu pour les dons des particuliers, autant de dispositions qui ont justifié la saisine pour avis de la commission des finances. La commission de la culture nous a d'ailleurs délégué au fond l'examen des articles 4, 5 et 5 . Avant d'aborder le détail du texte, permettez-moi de faire quelques remarques liminaires. Premièrement, ce texte confirme malheureusement, en creux, l'insuffisance des moyens budgétaires alloués à la préservation du patrimoine. L'État ne serait pas en mesure de faire face seul à la restauration de Notre-Dame de Paris. C'est d'ailleurs le mécénat qui finançait,

Troisièmement, ce texte révèle malheureusement une triple défiance : défiance à l'égard du ministère de la culture et des acteurs traditionnellement engagés dans la préservation du patrimoine

La commission des finances comme la commission de la culture ont mis en cohérence le projet de loi avec cette situation, d'autant qu'une telle structure aurait pour mérite de centraliser les financements et d'associer toutes les parties prenantes aux travaux de restauration de la cathédrale. Le choix de l'établissement public implique cependant de bien encadrer cette nouvelle structure, ce que nous allons faire. C'est dans cette optique que, conformément à l'engagement que j'ai pris devant la commission de la culture, j'ai déposé un amendement tendant à limiter sa durée à la période des travaux de restauration de la cathédrale postérieurs à l'incendie.

et l'établissement public afin d'assurer le respect de l'intention du donateur. Nous avons également prévu- c'est un point important -un versement progressif des fonds collectés en fonction de l'avancée des travaux et après transmission d'une estimation de la nature et des coûts de ceux-ci. Les fondations reconnues d'utilité publique ayant l'expérience de la gestion des dons, il faut se reposer sur elles. La commission des finances a également clarifié le dispositif prévu à l'article 4 relatif aux versements des collectivités territoriales, en précisant que ceux-ci devraient être considérés comme des dépenses d'investissement. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, mais il faut l'inscrire dans la loi.

monsieur le ministre, monsieur le rapporteur- je vous félicite pour votre travail sérieux et bienveillant, sauf sur un point essentiel, sur lequel nous reviendrons -, mes chers collègues, alors que Notre-Dame de Paris brûlait, même ceux qui voyaient les images en direct, si cruelles, ne voulaient et ne pouvaient y croire. n'était donc ni éternelle ni invincible. Tout était bien réel pourtant ; insupportable, mais réel. Nous nous sentions impuissants. Les pompiers, eux, agissaient avec héroïsme, faisaient ce qu'ils savent et doivent faire, avec professionnalisme et avec un immense courage.

On a tout dit ensuite de l'émotion partagée dans le monde entier et du formidable élan de solidarité qui a suivi. Les dons n'ont attendu aucun ordre ni aucune date de départ pour affluer. L'unanimité républicaine fut tout de suite au rendez-vous. Oui, il s'agissait de notre histoire, universelle, gravée dans le beau et dans la pierre, tant et si bien que notre pays, en guise d'hommage, plaça l'auteur des en tête des ventes de livres durant de nombreuses semaines après l'incendie. En communiant avec Victor Hugo, les Français montraient que Notre-Dame est de Paris, mais qu'elle appartient à toute la France et qu'elle vit dans le coeur et dans les yeux du monde entier. Oui, nous débattons aujourd'hui d'une grande cause culturelle, car il s'agit de création, d'architecture, de patrimoine historique.

mais pas pour faire une loi d'exception ! Tout ce qui est attentatoire à notre droit et à nos codes patiemment construits pour préserver les règles d'urbanisme, protéger l'environnement et, bien entendu, notre patrimoine doit être écarté. Nous connaissons tous les contraintes, les procédures parfois tatillonnes et les délais qui peuvent s'éterniser.

Mais enfin, ou l'État juge ses règles et ses codes mauvais, auquel cas il propose d'en changer, ou ils les trouvent bons et il nous propose de les respecter. Il y va de l'autorité de l'État et du ministère de la culture dans les prochaines années, pour chaque aménagement, chaque construction, chaque reconstruction, chaque restauration.

le bas, pour le culte et les visites, et même, et tel est notre souhait, de créer à l'extérieur un véritable musée-atelier des oeuvres et de la reconstruction de Notre-Dame. Pour cela, il faut que des moyens soient donnés, avec la Ville de Paris, pour que les abords soient compris dans la reconstruction. cinq ans pour que Notre-Dame soit sécurisée, rouverte et pour qu'on puisse la visiter, c'est possible. En revanche, il n'est pas sérieux de dire que le chantier serait achevé dans son ensemble d'ici à cinq ans, comme l'a réaffirmé le Président de la République vendredi.

La culture a passé l'âge du bon vouloir du Prince, pour devenir démocratique

l'incendie survenu le 15 avril dernier au sein de la cathédrale de Paris a suscité une forte émotion. Celle-ci témoigne du profond attachement de chacun à la richesse du patrimoine français, dont Notre-Dame est l'un des éléments les plus remarquables. Au travers de cette émotion, l'exécutif semble avoir perçu une attente, celle que soient le plus rapidement possible effacées les traces de ce sinistre, dont les conséquences auraient pu être beaucoup plus destructrices sans le professionnalisme et la célérité des pompiers parisiens. Dès le 16 avril, le Président de la République a souhaité s'exprimer dans le cadre d'une allocution télévisée. Alors qu'aucun diagnostic n'est établi, que l'intégrité des murs de l'édifice n'est pas encore totalement assurée, le chef de l'État déclare sa volonté de voir la restauration du monument achevée d'ici à cinq années. Pierre Dac disait que rien ne sert de courir si l'on n'est pas pressé. En effet, l'immédiateté, pour laquelle notre époque a un goût peut-être trop prononcé, n'est pas nécessairement un gage de bonne gouvernance. Si certaines situations appellent des réponses rapides, le chantier qui va s'ouvrir sur l'île de la Cité ne justifie aucun empressement particulier de notre part. Cette opinion est partagée par la quasi-totalité des groupes politiques du Sénat, qui ont porté des amendements de suppression de l'article 9 lors de l'examen du projet de loi en commission. Toutes dérogations ou adaptations s'appliquant aux règles d'urbanisme, de protection de l'environnement, de voirie et de transport, ainsi qu'aux règles de commande et de domanialité publiques, nous apparaissent très inopportunes. Un tel biais créerait un précédent dangereux en matière de restauration. Aucune contrainte temporelle ne s'impose en outre à nous, en tout cas aucune contrainte qui ait été portée à notre connaissance. Si le Gouvernement dispose d'éléments que nous ignorons, nous serions heureux qu'il les évoque au cours de notre débat. Quant au débat sur une possible évolution architecturale de l'édifice, nous estimons qu'il n'est pas de nature parlementaire. Même si nous sommes profondément attachés à la silhouette de cet édifice et de sa flèche, indissociable du coeur historique de Paris, nous gardons à l'esprit que le site de Notre-Dame s'est inscrit dans un continuum tout au long de son histoire, des Romains jusqu'à nos jours. Nous savons également à quel point ce type de débat, portant sur l'évolution d'un édifice d'une si grande notoriété, peut-être clivant au sein de la société. ans, lorsqu'il a été question d'implanter une pyramide de verre au sein de la cour du plus grand palais d'Europe, également témoin de 800 ans d'histoire, le débat fut âpre- degré zéro de l'architecture », on lança un « appel à l'insurrection » -, mais le résultat final a convaincu plus d'un sceptique. Aussi, je pense qu'il ne nous revient pas de nous prononcer sur ce point, sur lequel notre opinion compte après tout autant que celle de chaque Français.

le relèvement à 75 % du taux des déductions fiscales octroyées aux particuliers jusqu'à 1 000 euros ne nous paraît pas se justifier. Tout d'abord, ce taux représente encore un régime d'exception. Même si nous ne sommes pas arrivés au terme de la souscription et que nous ne connaissons pas l'estimation du coût de la restauration à venir, les projections laissent à penser que les fonds collectés seront suffisants. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'essayer de stimuler un élan qui est déjà remarquable par son ampleur. Ensuite, nous sommes favorables, dans un souci d'équité fiscale, à la proposition de M. Éblé de créer un crédit d'impôt afin que l'État puisse accompagner chaque Français, imposable ou non, dans cet effort. Il ne nous semble pas cohérent, d'un côté, de repousser cette proposition, en arguant de son coût pour l'État, comme l'a fait le Gouvernement à l'Assemblée nationale, et, de l'autre, de majorer une déduction d'impôt qui représentera, au bout du compte, également un coût supplémentaire pour l'État. Aussi, nous demanderons le maintien du taux de déduction de 66 %. Nous sommes conscients que le Premier ministre a rapidement proposé un taux de 75 % et que, jusqu'à présent, les donateurs ont effectué leur démarche en ayant à l'esprit ce cadre cadre élargi, mais nous connaissons aussi les difficultés budgétaires actuelles de l'État et leurs conséquences sur la vie quotidienne des Français. Si ce taux majoré n'a pas de pertinence, si ce n'est celle de venir grossir un catalogue de mesures d'exception, nous n'y souscrirons pas. Le Président de la République, dès le lendemain du sinistre, a appelé à l'union nationale, suspendant la restitution des conclusions du grand débat qu'il avait lancé.

que cette harmonie va se poursuivre au cours de notre débat aujourd'hui. Il est essentiel, si le Sénat s'accorde une nouvelle fois sur une proposition rassemblant le plus grand nombre d'entre nous, que les discussions avec nos collègues députés sur une rédaction commune soient animées du même esprit. La renaissance de Notre-Dame n'a pas de marqueur politique. L'unité que le chef de l'État a appelée de ses voeux à la suite de ce sinistre doit aussi se traduire par une vision commune à l'ensemble de la représentation nationale.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes très chers collègues : « J'ai voté contre le projet de loi sur la restauration de Notre-Dame de Paris, car la loi en question est à la fois inutile et toxique, dans la mesure où, au nom d'une urgence imaginaire, elle remet en cause toutes les garanties procédurales et parlementaires visant à la préservation du patrimoine et de l'environnement. » Ces propos très sévères à l'endroit du texte que vous venez de nous présenter, monsieur le ministre, émanent non pas de votre opposition, mais de Jean-Louis Bourlanges, un parlementaire aguerri de votre majorité à l'Assemblée nationale. Comme cet ancien collègue de ma région, pour lequel j'ai beaucoup de considération, et bien d'autres, je ne pense pas que les Français souhaitent que l'on malmène l'État de droit. Le Gouvernement a fait le choix de répondre à l'événement exceptionnel qu'a constitué cet incendie par le dépôt immédiat d'un projet de loi de dérogations : dérogations au code de l'urbanisme et de l'environnement, au code des marchés publics et au code du patrimoine. Cela donne le sentiment que notre pays ne disposerait ni de l'organisation, ni de l'expertise, ni des outils pour faire face à un chantier d'une telle dimension. Je comprends mal la défiance qui transparaît dans la plupart des dispositions de ce texte à l'égard de la capacité du ministère de la culture à assumer ce chantier de restauration. Sans la qualité et l'engagement quotidien de ses personnels, sans la formation dispensée au sein des écoles placées sous sa tutelle, la réputation de notre pays dans ce domaine ne serait pas la même. Nous avons vu avec quelle réactivité les équipes du ministère, de la DRAC et de la Ville de Paris sont intervenues pour mettre à l'abri les oeuvres de la cathédrale. Elles sont à pied d'oeuvre depuis le 15 avril pour parer à la situation d'urgence impérieuse. Nous voulons ici leur rendre hommage, ainsi bien sûr qu'aux pompiers, qui ont empêché le pire. Que vous vouliez aller vite, pourquoi pas, au regard de l'émotion qu'a suscitée ce sinistre et de la nécessité de mobiliser autour de ce chantier ; à condition que cela reste un objectif et non pas un impératif. Je constate que, grâce à la générosité de très nombreux donateurs, nous aurons la chance de disposer de fonds considérables, qui permettront d'avancer vite. Mais s'il est important, l'argent ne fait pas tout. Il faut en effet effectuer un énorme travail de déblaiement, de dépollution, de sécurisation et de diagnostic, auquel se sont déjà attelées les équipes. À cet égard, il faudrait méditer cette phrase de l'auteur de, Victor Hugo, « Le temps est l'architecte et le peuple est maçon », pour comprendre que nous ne sommes, artisans comme décideurs, qu'un des petits maillons de la chaîne de l'histoire de la construction et de la restauration des cathédrales. Il en va ainsi depuis le Moyen Âge ! J'insiste, monsieur le ministre, car on ne peut ignorer ce qui constitue le socle de notre système de protection du patrimoine. Difficile au Sénat de ne pas penser au rôle joué au XIX siècle par Prosper Mérimée, celui-là même qui confia le chantier de Notre-Dame de Paris en 1843 à Viollet-le-Duc lorsqu'il occupait les fonctions d'inspecteur général des monuments historiques. Son action trouva son aboutissement en 1913 avec la loi sur les monuments historiques, dont de nombreuses dispositions sont encore aujourd'hui en vigueur et ont été modernisées et approfondies, il y a trois ans, dans le cadre de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Je rappelle que Prosper Mérimée a été sénateur

Comment garantir ensuite le respect de ces règles par les autres propriétaires de monuments historiques si celui qui les édicte, l'État, s'en affranchit pour mener l'un des chantiers les plus emblématiques de France ? Comment comprendre, s'agissant de l'application du code des marchés publics, qu'il puisse y avoir deux poids deux mesures ? Oui, ce chantier doit être exemplaire, par respect pour toutes celles et tous ceux qui ont partagé une même et profonde émotion, pour les donateurs aussi, petits et grands, qui ont répondu massivement à l'appel de la souscription. Je veux rappeler que Notre-Dame a constitué un élément déterminant pour justifier l'inscription, en 1991, du site « Paris, rives de la Seine » au patrimoine mondial de l'Unesco. Il est très étonnant que ce classement n'ait pas été pris en compte dans le projet de loi, sans doute par précipitation. Je remercie donc le rapporteur d'avoir corrigé cet oubli et rappelé ses implications. Notre législation, particulièrement complète et protectrice, a été jusqu'ici mise en avant par les autorités auprès de l'Unesco afin de garantir que la valeur universelle exceptionnelle de « Rives de la Seine » serait correctement protégée. Suspendre l'application d'un certain nombre de dispositions

Personnellement, je crois que, globalement, les Français veulent retrouver leur cathédrale, la silhouette familière de sa flèche dans le ciel de Paris. S'il n'appartient pas au législateur de définir les choix architecturaux ou techniques, il lui revient de rappeler les obligations d'en préserver l'« authenticité » et l'« intégrité » : tels sont les termes figurant dans les textes en vigueur. Cela signifie aussi qu'il faut prendre en compte l'inscription de Notre-Dame dans un paysage urbain préexistant, défini, qui inclut un certain nombre d'édifices à remettre en perspective, dont la Sainte-Chapelle. Je veux insister sur le rôle essentiel et pivot de l'architecte en chef du monument, Philippe Villeneuve, et de son équipe, sous l'égide duquel toute décision devra être prise. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, présidée par notre excellent collègue Jean-Pierre Leleux, doit par ailleurs être étroitement associée à ce chantier, du début à la fin. Enfin, nous pensons que le chantier doit aussi être une occasion de valoriser les métiers du patrimoine, dont plusieurs sont menacés, faute de vocations, même s'il n'y a pas aujourd'hui de risque de pénurie sur le chantier.

Ces métiers ont de l'avenir, à condition que l'on veille précisément à ce que les délais de réalisation du chantier ne viennent pas déstabiliser une filière dont le rôle pour l'économie de nos territoires ne doit pas être négligé. Ce secteur est constitué de petites entreprises qui se trouveraient, de fait, écartées si des dérogations permettaient de recourir à des marchés globaux au lieu d'allotir le chantier. Il faut aussi articuler le chantier de Notre-Dame avec les autres chantiers de restauration, en cours ou planifiés sur le territoire de l'Hexagone, pour ne pas priver ces derniers de la main-d'oeuvre nécessaire.

Je n'ai pu aborder, hélas ! au nom du groupe Union Centriste, tous les aspects de ce texte, mais nous faisons confiance aux deux rapporteurs. Qu'ils soient sincèrement chaleureusement remerciés, car les délais qu'ils ont eus pour travailler étaient complètement fous. De la même manière, je salue l'ensemble de mes collègues de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui, en dépit des délais impartis, se sont considérablement impliqués, de jour comme de nuit, ces sept dernières

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous tous, j'ai été profondément touché par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, incendie qui l'a lourdement dégradée, mais heureusement pas détruite. J'étais sur le pont des Arts

pour appartenir au patrimoine mondial. La date du 15 avril restera sans doute gravée dans les mémoires, du fait de l'ampleur de l'incendie, mais également, cela a été dit, du courage des soldats du feu, de tous les hommes de sécurité qui ont réussi à sauver non seulement l'édifice, mais les éléments qu'il contenait. Cette date restera également marquée par l'élan de solidarité qui a suivi, de nombreux Français ou étrangers, des entreprises, des collectivités, des citoyens sans fortune ou disposant au contraire d'une grande fortune s'étant mobilisés pour offrir quelques euros, qui des sommes bien plus importantes. Notre-Dame appartient bien à notre patrimoine historique, spirituel, architectural, littéraire. Sa restauration doit répondre à de multiples attentes. Elle doit être à la hauteur de cet élan de soutien massif. Même si, aux dires de certains, ce projet de loi n'était pas indispensable, il a le mérite de nous permettre d'échanger sur des sujets qui forment notre société : la solidarité et la conception que nous nous faisons de la préservation de notre patrimoine. Le mécénat constitue un puissant levier pour agir à l'échelon local en faveur de l'intérêt général. Les Français sont attachés à leur patrimoine, à leurs 42 300 monuments historiques répartis sur l'ensemble du territoire, mais mais également à l'ensemble du petit patrimoine monumental, cultuel ou vernaculaire. Pourtant, les acteurs de proximité, notamment les collectivités territoriales, sont parfois loin de s'être approprié sa protection.

de refonder le lien entre l'État et les contribuables, sur la base de l'intérêt général, tout en favorisant l'initiative privée. Cela nous conduit évidemment à nous interroger également sur la restauration que nous souhaitons pour Notre-Dame. Victor Hugo écrivait : « Chaque flot du temps superpose son alluvion, chaque race dépose sa couche sur le monument, chaque individu apporte sa pierre. » Il avait raison. Même si nous devons veiller à préserver l'identité, l'authenticité et l'intégrité du monument, ne nous empêchons pas de faire preuve d'audace et de laisser nos générations marquer cet édifice de leur empreinte, comme cela s'est fait au fil des siècles, à de nombreuses reprises. Pourquoi nous en priverions-nous ? Le projet de loi permet à la fois d'encadrer cet élan de générosité sans précédent et de préparer au mieux les mois et les années à venir pour la conservation et la restauration de notre chère cathédrale. Les articles 1 à 5 vont ainsi dans le bon sens. Ils permettent d'éviter toute incertitude quant à l'utilisation des fonds, aux possibilités de collectes et à la gestion des versements. Le texte permettra d'organiser la souscription dans un cadre sécurisé et transparent, en faisant appel aux acteurs de référence en matière de levées de fonds et de philanthropie.

Cette exemplarité devra aussi s'appliquer tout au long de la préparation du chantier, puis lors de la réalisation des travaux. Il sera également essentiel de prendre en compte les différents usages cultuels, culturels et touristiques de Notre-Dame pour que sa restauration permette d'améliorer le fonctionnement quotidien. N'oublions pas l'hyperfréquentation dont sont souvent victimes les sites monumentaux. La création d'un établissement à caractère administratif de l'État semble pertinente, compte tenu de la nature exceptionnelle du chantier et de la nécessité de réunir toutes les parties prenantes.

du domaine de la loi ? La France est une terre de patrimoine. La propriété de ce patrimoine est souvent publique, parfois privée. Tous les propriétaires, qu'il s'agisse de collectivités ou de personnes privées, n'ont pas, dans la plupart des cas,

S'agissant de Notre-Dame, le Gouvernement a souhaité que l'immense chantier de sa reconstruction, de sa restauration soit exempt de cette réglementation, à la fois parce que les plus grands experts sont déjà à l'oeuvre pour organiser la restauration, mais aussi pour gagner le temps nécessaire à opérer ces travaux dans des délais raisonnables. Je vais sans doute vous choquer,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en préalable à mon propos, je tiens tout d'abord à saluer ici l'esprit de cohésion et de solidarité nationale qui a présidé le soir du 15 avril lorsque nous avons appris l'incendie qui a très lourdement endommagé ce joyau national qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Chacun a justement souligné l'extraordinaire réactivité de nos soldats du feu, les risques considérables qu'ils ont pris pour sauver ce qui pouvait encore l'être et le « sans-faute » du commandement des opérations, qui, dans l'urgence de ce funeste moment, a mis en oeuvre les meilleurs choix qui pouvaient être pris en pareille situation. Je le dis ici : l'opération « Sauver Notre-Dame » restera dans l'histoire comme un exemple de bravoure et d'intelligence en matière d'opération de sécurité civile, et ce à l'échelle mondiale ! Je veux saluer aussi l'extrême réactivité du Président de la République, quelques dizaines de minutes seulement après le déclenchement de l'incendie, a choisi d'annuler l'intervention télévisée très attendue qu'il devait faire pour se rendre immédiatement sur les lieux du sinistre et valider les décisions qui étaient à prendre en temps réel. C'est avec le même esprit de détermination que le Président a décidé très rapidement d'engager « l'après-incendie » et que le Gouvernement a présenté un texte de loi pour conserver et restaurer Notre-Dame, pour réparer cette plaie ouverte laissée au coeur de Paris, au coeur de la France et au coeur de chacune et de chacun d'entre nous. Non, Paris n'est pas Rome, et le culte magnifié des ruines n'appartient pas à notre culture, n'en déplaise à quelques esprits romantiques. L'amour de notre patrimoine, depuis plusieurs siècles, nous a toujours conduits à le protéger, à l'entretenir, à le faire vivre ou revivre. Il faut le rappeler ici : aucun pays au monde ne prête autant d'attention que le nôtre à son patrimoine. Alors, pour ce faire, l'argent manque toujours, mais ce manque doit être mis en regard de l'incroyable richesse de notre patrimoine, qui ne cesse, siècle après siècle, décennie après décennie, de s'étoffer. Depuis ce drame, et surtout depuis les polémiques attisées par certains, on entend sur ces bancs un cortège de lamentations et de dénonciations quant au manquement dont l'État serait coupable à l'endroit de notre patrimoine national. disent que ce serait l'actuel Gouvernement, celui qui précisément a engagé le plus d'actions en faveur du patrimoine au cours des trente dernières années, qui serait le coupable tout désigné de ce prétendu abandon. Je rappelle tout de même que Notre-Dame de Paris n'était pas en déshérence au moment du drame et que le terrible incendie s'est précisément produit durant l'important chantier de rénovation de sa flèche. Je rappelle aussi que lors du dernier projet de loi de finances, discuté en fin d'année passée au Sénat, le président de notre commission des finances, Vincent Éblé, très fin connaisseur du patrimoine, donnait même un satisfecit à l'accroissement des engagements financiers de l'État dans ce domaine. Je rappelle encore que, toujours lors de ce même projet de loi de finances, et à l'exception d'un amendement assez général du groupe CRCE, aucun amendement visant à accroître davantage ces budgets n'a été déposé dans notre chambre. Mais venons-en au fond du sujet, c'est-à-dire au texte de loi tel que profondément amendé en commission, la semaine dernière, et que nous étudions aujourd'hui. La commission a bien entendu le droit de récrire la proposition initiale si celle-ci ne lui convient pas. dans le cas présent, je cherche encore la cohérence et la sincérité effective du propos. En commission, le président Bruno Retailleau a solennellement dénoncé l'ombre projetée de l'« hybris présidentielle » dans ce dossier, affirmant même au passage qu'il n'y avait nul besoin d'une loi pour restaurer Notre-Dame. Franchement, je dois dire qu'on trouve bien pire exemple d'hybris présidentielle sous la V République, y compris chez certains ex ou futurs candidats à la fonction. D'ailleurs, il est intéressant aussi de noter que nos collègues Les Républicains au Sénat, contrairement à leurs homologues de l'Assemblée nationale, ont fait preuve de retenue en ne déposant aucun amendement de suppression de l'alinéa 2 de l'article 1, qui place pourtant la souscription ouverte « sous la haute autorité du Président de la République française ». Je ne reviendrai pas ici point par point sur les différents ajouts et amputations auxquels notre commission s'est livrée. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'étude du texte. Je voudrais, dans le temps qui me reste, simplement revenir sur l'un des points qui semble cristalliser la polémique : il s'agit de la fameuse question de l'authenticité et de la reconstruction à l'identique de l'édifice. Je veux souligner ici le procédé pour le moins étonnant, pour ne pas dire fallacieux, qui a présidé à la réécriture de l'alinéa 2 de l'article 2. Pour arguer en faveur d'une reconstruction à l'identique de la cathédrale et la restituer « dans le dernier état visuel connu », le rapporteur n'hésite à invoquer la Charte de Venise de 1964, qui n'a aucune valeur contraignante et qui, par ailleurs, a fait l'objet d'une intense rediscussion pour être modifiée par le Document de Nara de 1994 sur l'authenticité et l'interprétation relative à lui donner. L'invocation dans ce même alinéa de la Convention de l'Unesco de 1972 sur le patrimoine mondial, qui elle est contraignante, est néanmoins inappropriée puisque dans aucun de ses articles il n'est fait mention d'une obligation de respecter une quelconque authenticité ou intégrité des monuments

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans son, Grégoire de Tours rapporte que de son temps, en 586, l'île de la Cité fut dévastée par un terrible incendie. L'historien explique que la consécration de la ville la protégeait jadis contre le désastre des flammes, mais que lors du curage des égouts « on y avait trouvé un serpent et un loir d'airain ; qu'après qu'on les eut ôtés il parut dans Paris des loirs et des serpents sans nombre, et qu'après cela la ville fut prise de l'incendie ». Aussi loin que nous portent dans le temps les écrits et les témoignages matériels des humains, l'île de la Cité est l'espace des destructions, des relèvements et des créations. La cathédrale de Notre-Dame a succédé ainsi à un groupe épiscopal plus ancien qui fut détruit et dont les pierres ont été réutilisées pour l'édifice nouveau. Enfin, la configuration actuelle des lieux doit beaucoup aux travaux de Rambuteau, de Viollet-le-Duc et surtout d'Haussmann. Sans le dévouement exceptionnel des pompiers, des personnels du ministère de la culture et de la mairie de Paris, du diocèse et des entreprises, il est possible que la vieille cathédrale eût connu un destin aussi funeste que les édifices qui la précédèrent. Aujourd'hui, l'essentiel est sauvé, mais la très longue histoire du bâtiment et du lieu nous impose l'humilité. En juillet 1798, le général Bonaparte, devant les pyramides, déclarait : « Songez que du haut de ces monuments quarante siècles vous contemplent. Regardant Notre-Dame, nous pourrions dire à sa suite : du haut de ces deux tours vingt siècles nous regardent. Non seulement il convient d'agir en pleine connaissance de la richesse patrimoniale de ce monument et de son environnement architectural, mais nous devons aussi intervenir dans le respect de sa destination première et actuelle, celle d'un lieu de culte qui tente d'offrir à ses pratiquants un espace de recueillement dans un bâtiment qui est le plus visité d'une capitale qui est la première destination touristique mondiale. Le ministère de la culture et ses services patrimoniaux ont une pratique longue et assurée de la gestion de ces problématiques multiples, car celles-ci sont consubstantielles de la plupart des travaux réalisés dans des monuments historiques. Certes, il est heureusement rare qu'un tel sinistre survienne dans un ensemble architectural aussi vaste et complexe que celui de la cathédrale Notre-Dame. les lois et règlements forgés à la suite d'une expérience pluriséculaire dans ce domaine offrent justement les cadres adaptés pour élaborer, discuter et mettre en oeuvre les projets de restauration les plus difficiles. Fort de ces expériences anciennes, notre pays a contribué à l'élaboration d'une doctrine qui a servi de socle aux traités internationaux destinés à protéger le patrimoine historique : la Charte de Venise, la Convention de Malte et le Document de Nara. À propos du concept d'authenticité introduit par la Charte de Venise, ce dernier texte précise : « Les couches d'histoire acquises au fil du temps par un bien culturel sont considérées comme des attributs authentiques de ce bien culturel. Tous ces travaux ont contribué à la constitution d'une conscience patrimoniale internationale qui a pour dessein « de clarifier et d'éclairer la mémoire collective de l'humanité Elle s'est manifestée avec force lors de la destruction des Bouddhas de Bâmiyân en Afghanistan, ou des vestiges archéologiques de Palmyre en Syrie. Par un renversement singulier du destin, cette conscience patrimoniale universelle s'est exprimée, dès le 15 avril, pour nous témoigner sa tristesse, sa compassion et sa volonté de participer à nos côtés au relèvement de ce qui a été détruit. Cette mansuétude universelle nous honore et nous oblige. Elle doit nous astreindre à respecter scrupuleusement les préconisations patrimoniales des chartes internationales pour l'élaboration desquelles notre pays a fortement collaboré. La très récente loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine peut être considérée comme une transposition aboutie dans le droit français de ces principes. Nous ne comprenons donc pas pourquoi vous nous proposez d'y déroger aujourd'hui. Certes, le chantier de restauration de la cathédrale sera exceptionnel par sa durée et les moyens humains et financiers qui seront mobilisés, mais rien dans son organisation juridique et administrative ne justifie cette loi d'exception. S'agissant de l'article 8 et de votre souhait d'instituer par ordonnance un nouvel établissement public chargé de la rénovation, dans l'étude d'impact qui accompagne ce projet de loi, le Gouvernement défend son utilité par la seule nécessité d'assurer une gouvernance du chantier « reflétant pleinement la diversité des personnes intéressées à la restauration ». Est-ce à dire qu'avant l'incendie la collaboration entre le ministère de la culture et ses services, la mairie de Paris et le diocèse était déficiente ? Le sentiment qui prévaut est plutôt celui d'une dépossession des autorités actuellement compétentes au profit d'un dispositif contrôlé depuis le plus haut sommet de l'État. Sur le fond, cet exercice de contournement de la loi et des services chargés de l'appliquer jette le discrédit sur toutes nos institutions patrimoniales pour organiser le fait du Prince. Comment obtenir de l'élu et du citoyen le respect de la loi si le premier magistrat de la République exige de nous, par ce texte, de s'en affranchir absolument ? La parole

nous sortons d'une séquence électorale qui a mis en lumière nos différences. Mais s'il est des moments dans notre vie commune qui peuvent nous opposer, il en est d'autres qui nous rassemblent parce qu'ils transcendent nos désaccords, et l'incendie dramatique de Notre-Dame de Paris a été évidemment de ceux-là. Ce soir-là, le feu a éteint pour un temps nos querelles, et tous nous étions derrière ceux qui s'élançaient au coeur du brasier, ces pompiers au courage exemplaire. Ce soir-là, les fumées s'échappant de Notre-Dame ont pour un instant recouvert les clivages et rallié les regards de tous ces Français reliés dans une même émotion et rassemblés comme une seule nation. Ce soir-là sous les flammes, mes chers collègues, a percé notre âme, celle d'un peuple qui, malgré ses fractures, ses blessures, a montré qu'il pouvait encore vivre du même esprit, celui de l'unité, aimer du même coeur, un coeur souffrant tant les maux qui divisent la France font souffrir les Français, mais un coeur toujours battant pour ce qui nous rassemble. Et d'un mal peut sortir un bien. Ce soir-là, du malheur a surgi, comme un bonheur, notre bien le plus précieux, le plus fragile aussi : l'unité nationale, cette grande oeuvre française, qui toujours est à recommencer. Il y a là comme un signe réconfortant. je crains que ce signe ne soit obscurci par le signal que vous envoyez avec certaines dispositions de ce projet de loi, un projet qui me semble à contretemps, car Notre-Dame de Paris est d'abord l'oeuvre du temps. Il a fallu des siècles pour écrire « ce livre d'histoire de France » dont parle Jules Michelet, des siècles de patience pour conjuguer ses formes, du choeur jusqu'aux portails, des siècles de persévérance pour ciseler cette synthèse de roses, de stalles et de chimères. Or à la patience vous substituez l'urgence, qui justifierait de s'exonérer de toutes les règles urbanistiques, patrimoniales du code des marchés publics ; et à la persévérance vous substituez la performance : reconstruire Notre-Dame en cinq ans Alors, y a-t-il urgence ? Oui, il y a une urgence à sécuriser, à consolider, à protéger, en liaison étroite avec les acteurs culturels, mais aussi, comme vient de le dire Pierre Ouzoulias,

Et même s'il faut d'urgence protéger l'édifice, il n'y a rien qui justifie de restaurer dans l'urgence, à la va-vite. Faudrait-il bâcler le chantier pour boucler un calendrier ? Choisir le béton plutôt que le chêne pour une charpente qu'après tout le flot de touristes n'apercevra même pas ? Faudrait-il restaurer ce haut lieu de notre identité comme on construit ces non-lieux de notre surmodernité : au plus simple, au plus vite parce que le présent n'attend pas, exige son dû, et peu importe le don du passé ? Non, Notre-Dame mérite plus, Notre-Dame mérite mieux ! Elle mérite plus que ce « présentisme » dans lequel vous vous enfermez. Elle mérite mieux que ce « bougisme » auquel, une fois de plus, vous cédez. Car cette urgence, c'est vous qui l'avez créée, comme l'a d'ailleurs souligné avec intelligence Jean-Louis Bourlanges, qui appartient à votre propre majorité. En la créant, vous prenez le risque de décrédibiliser l'État qui, avec l'article 9 de ce

c'est pour vous ; l'exception, c'est pour nous. » Très bien ! Une fois de plus, l'État ne montre pas l'exemple. Et quel contre-exemple ! Pour Notre-Dame de Paris, de deux choses l'une : soit ces règles sont mauvaises, et dans ce cas ne vous en exonérez pas, mais supprimez-les supprimez-les pour tout le monde ; ... Bien sûr ! ... soit elles sont utiles et nécessaires, ce que je pense, et alors respectez-les ! Plus grave encore, vous prenez le risque de décrédibiliser la France : parce que c'est sous son impulsion que l'Unesco a établi des critères précis pour la protection du patrimoine mondial de l'humanité, parce que c'est aussi grâce à la France que la Charte de Venise a été adoptée, et parce qu'enfin c'est en France que l'on trouve une excellence inégalée, celle de nos architectes en chef, de nos historiens de l'art, celle aussi de nos compagnons. Leur savoir-faire est mondialement reconnu, alors accordez-leur accordez-leur un peu de crédit quand ils vous exhortent à vous accorder un peu de temps ; accordez-leur un peu de considération en leur confiant, à eux plutôt qu'à d'éventuels gagnants d'un concours international, la reconstruction de la flèche de Viollet-le-Duc. Quant à la performance, vouloir reconstruire Notre-Dame « plus belle encore », pour reprendre les mots du Président de la République, c'est, pardonnez-moi, faire preuve d'une ambition qui confine à la prétention.

la prouesse d'un chef d'État qui voudrait laisser sa marque au-dessus de Notre-Dame de Paris. La seule marque que nos compatriotes veulent voir, celle à laquelle ils sont réellement attachés, ce n'est pas celle d'un Président, c'est la marque du temps, la trace du génie des siècles inscrite dans la pierre de Notre-Dame. De même, le seul geste que nos concitoyens attendent, ce n'est pas un geste de « modernité », comme cet improbable « geste architectural contemporain » voulu par Emmanuel Macron, mais c'est un geste de fidélité, geste de fidélité, qui a quelque chose à voir avec tous ces gestes de générosité dont ont fait preuve des milliers de Français. Car pourquoi ont-ils donné

les préférences esthétiques importent peu : il s'agit non pas de préférer, mais de respecter ; il s'agit non pas de « disrupter », mais de restaurer. Du reste, le seul vrai juge en matière d'art, c'est le temps. C'est dans la profondeur du temps que naît la grandeur des oeuvres. Notre-Dame de Paris est née voilà neuf siècles. Le temps a fait de ce joyau français un trésor d'humanité. Alors, si vous voulez redonner tout son éclat à ce trésor,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, oui, Notre-Dame est exceptionnelle, mais elle ne doit pas faite l'objet d'une loi d'exception. L'incendie n'a pas uniquement ravivé notre émotion, il a aussi réveillé notre conscience collective sur la place éminente du monument dans notre histoire et dans notre présent. Notre-Dame nous était familière, tellement familière que nous avions fini par oublier qu'elle était vulnérable. Parce qu'elle est là depuis des siècles, ayant franchi des époques parfois tumultueuses, nous étions enfermés dans la certitude de son immobilité, comme le dit l'historien Yann Potin. En bref, le temps passe, mais Notre-Dame reste. C'est pourquoi, le 15 avril dernier, nous avons tous été abasourdis : nous avons redécouvert que Notre-Dame était fragile. Les élans d'affection spontanés, mêlés d'une profonde inquiétude sur la survivance de l'édifice, ont soudainement mis en lumière l'attachement viscéral des Français, mais également du monde entier, à cette cathédrale qui, depuis fort longtemps, était devenue bien plus que cela. Partie intégrante du site « Paris, rives de la Seine », inscrit au patrimoine mondial, Notre-Dame est une évidence : elle est un bien commun, pas seulement national, mais de l'humanité tout entière. À l'heure de sa restauration, cette vérité nous oblige. En tant que législateurs, le cadre et les lignes directrices que nous allons fixer conditionneront en partie la fluidité et la réussite du projet. C'est donc une réelle responsabilité qui nous incombe, responsabilité dont nous allons débattre aujourd'hui, mais qui a en réalité une portée internationale. Au-delà du financement du projet, le premier facteur décisif se situe au niveau de la gouvernance du futur établissement qui conduira et coordonnera les opérations de restauration. Sur ce point, nous ne pouvons que saluer le travail du rapporteur et les avancées obtenues dès le stade de la commission, puisqu'il est désormais précisé qu'il s'agira d'un établissement public à caractère administratif- EPA -de l'État placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Pour notre part, nous souhaiterions encore affiner et clarifier ce schéma, en inscrivant un principe simple dans la loi : la séparation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre. Si l'EPA a la charge de la maîtrise d'ouvrage, les opérations de maîtrise d'oeuvre doivent bien sûr être conduites sous la direction d'un architecte en chef des monuments historiques. Ce qui est en jeu autour de ces considérations d'apparence technique, c'est bien la qualité de la restauration de Notre-Dame. Or qui mieux que les services du patrimoine du ministère de la culture, reconnus pour leur expérience et leur expertise, sont-ils à même d'assurer cette qualité ? Architectes, inspecteurs, conservateurs, tous sont qualifiés, compétents et ont fait leurs preuves pour réussir un tel chantier faisons-leur confiance ! En revanche, ils ne peuvent pas tout, et ils ne peuvent pas aller à l'encontre des règles qui auront été définies par la loi. C'est pour cette raison qu'en préambule de mon intervention j'ai clairement exprimé mon opposition à une loi d'exception. Le message de la commission a été limpide, monsieur le ministre : nous vous soutenons pleinement, mais nous ne voulons aucunement d'une loi ÉLAN. Ainsi, nous ne voulons pas entendre parler de dérogations aux codes du patrimoine, de l'environnement, de l'urbanisme, de la commande publique. Nous ne voulons pas rebâtir « plus vite » Notre-Dame ; nous voulons « bien » la rebâtir. Elle mérite une restauration exemplaire, dans la transparence la plus totale, qui s'oppose radicalement à la logique de « dénormer » par ordonnances, et selon les règles de protection patrimoniale de droit commun saluées unanimement à travers le monde entier pour leur efficacité. Cet esprit soucieux du patrimoine, ce respect à l'égard de la pierre et du monument doivent être d'autant plus confirmés et affutés qu'il est question justement de Notre-Dame. Y déroger, c'est affaiblir considérablement et durablement la tradition de préservation patrimoniale de notre pays. Enfin, Notre-Dame n'est pas un lieu détaché ; elle est au coeur de la Cité, au kilomètre zéro de notre mémoire commune. Si beaucoup d'entre nous ont été affectés par l'incendie, c'est précisément parce que nous sommes nombreux à nous être approprié cette « dame aux multiples visages En un sens, l'histoire de Notre-Dame est une histoire d'appropriation perpétuelle et de symbolisme politique récurrent. Je crois qu'il est important que ce processus d'appropriation perdure pendant les travaux de restauration, autrement dit que Notre-Dame demeure ouverte sur la ville et sur le monde, notamment l'aménagement des abords, qui permettra d'organiser des ateliers, d'expliquer le chantier et, par conséquent, d'accueillir le public. D'ailleurs, cette période est de nature à valoriser, et peut-être même à redécouvrir, tous ces métiers du patrimoine qui travaillent les matériaux d'une main d'orfèvre.

» Monsieur le ministre, mes chers collègues, afin que ce « trait de lumière » redevienne éblouissant, prenons le temps qu'il faut. Le temps de Notre-Dame n'est pas le nôtre, et nul ne peut être plus grand ni plus rapide qu'une cathédrale

a submergé nos coeurs d'une émotion collective simultanée, dans une communion- osons le dire -jamais constatée dans l'histoire. Dans les minutes qui ont suivi, un extraordinaire élan de générosité se manifestait et les dons affluaient des quatre coins du monde. Cette « brûlure à l'âme » révélait- ou réveillait -cette perception intime de notre conscience profonde que Notre-Dame de Paris représentait plus qu'un monument historique traditionnel, mais aussi le symbole de notre civilisation européenne quelque peu enfoui au fond de nos mémoires. Il était légitime que le Président de la République, partageant cette émotion populaire unanime, s'exprimât rapidement. C'est- et l'on peut le comprendre -sous l'effet d'une forte émotion qu'il affirma : « Nous rebâtirons Notre-Dame, dans un délai de cinq ans, plus belle encore. Il n'en fallut pas plus pour que l'émotion, jusqu'alors consensuelle, se transformât en une polémique clivante sur les délais annoncés, le parti architectural qui allait présider à cette restauration, les risques d'un concours international pour reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc, l'idée d'un « geste architectural », les matériaux qui seraient utilisés, etc. Le Sénat, vous le savez, monsieur le ministre, a toujours manifesté une grande vigilance sur les sujets patrimoniaux, à la recherche d'un consensus sur toutes les travées, estimant que l'héritage commun que nous avons entre les mains devait échapper aux combats politiciens et partisans, le patrimoine légué par les générations qui nous ont précédés méritant respect, sérénité et humilité. C'est, une fois encore, ce que nous avons fait, attentifs au débat public, en nous référant à l'histoire exceptionnelle et universelle de ce vénérable monument et en le resituant dans son contexte paysager au coeur de Paris,

en tout point à l'exposé que vient de faire M. le rapporteur dans cette discussion générale. Je souhaite simplement insister sur trois éléments d'appréciation, plus personnels peut-être, qui marquent de façon plus volontariste encore mon souhait de voir restituer le monument de Notre-Dame dans un état le plus proche possible de celui dans lequel il était la veille du sinistre. Le premier point concerne la reconstruction dite « à l'identique ». Je mesure l'ambiguïté mais je souhaite, à l'instar d'une majorité d'historiens et de spécialistes du patrimoine, qu'elle soit respectée autant que possible. C'est la raison pour laquelle je demande, non seulement une « restitution visuelle », expression qui figure actuellement dans le texte, mais également une restitution respectueuse de l'état architectural antérieur au sinistre, y compris dans dans les matériaux utilisés. Nous avons une opportunité extraordinaire de valoriser les compétences et les savoir-faire exceptionnels de nos experts et artisans du patrimoine, une occasion unique d'organiser une opération d'envergure européenne qui permettra de transmettre ces savoir-faire, dans l'esprit du compagnonnage, et, ce faisant, de revaloriser le travail manuel noble, pour lequel nous commençons à manquer de vocations. Puis-je vous rappeler, monsieur le ministre, que vous avez déposé, au nom de la France, à l'Unesco, il y a tout juste deux mois, aux côtés de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Norvège et de la Suisse, une candidature au patrimoine culturel immatériel de l'humanité portant sur « les techniques artisanales et les pratiques coutumières des ateliers des cathédrales en Europe » Quant aux matériaux, il appartiendra au maître d'ouvrage de nous prouver que l'usage du bois, des pierres et même du plomb est incompatible avec les nécessités contemporaines. Nous disposons de l'ensemble des documents d'archives détaillant très précisément la disposition et l'agencement de tous les éléments constitutifs du monument à la date du sinistre. Le deuxième point concerne l'opérateur qui sera maître d'ouvrage délégué. Je ne comprends pas qu'il soit nécessaire de créer un opérateur dédié à la restitution de Notre-Dame. Cet opérateur existe déjà : il s'agit de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, l'Oppic, dont c'est précisément la mission. Ce dernier a opéré et opère encore sur d'importants chantiers touchant des monuments historiques majeurs, chantiers dans lesquels il a su démontrer son expérience et sa compétence. Et je ne vois pas pourquoi, au moment même où le Premier ministre demande que des opérateurs de l'État soient supprimés, nous en créerions un nouveau alors que nous avons ce qu'il faut.

J'ai tremblé, monsieur le ministre, quand j'ai entendu Mme Sibeth Ndiaye, porte-parole du Gouvernement, déclarer juste après la conférence de presse du Président de la République, que le but était « d'accélérer les travaux » Vous comprendrez, monsieur le ministre, combien ce type de déclarations, quand il s'agit de notre patrimoine, qui plus est de Notre-Dame de Paris, peut soulever de légitimes inquiétudes. que ces règles, notamment dans le domaine de la protection du patrimoine, ne sont nullement un frein à l'exécution des travaux, que tout l'arsenal réglementaire existe déjà dans nos textes, y compris la possibilité de raccourcir les délais, je me réjouis de la suppression de cet article 9 par la commission de la culture, sur proposition de notre collègue rapporteur Alain Schmitz. Je reviendrai sur ces points lors de l'examen des articles, mais je pense

La séance est reprise.

y compris sur nos travées au Sénat, vous l'avez compris, à vouloir aussi que le monument garde à terme son allure, son profil et retrouve sa silhouette si familière. Par ailleurs, le principe d'égalité appelle le législateur à un respect scrupuleux

mais pour tous et sur tout le territoire ! Dans le cas contraire, il faut faire avec l'existant. C'est possible, qu'il s'agisse de la création d'un établissement public, des déductions fiscales ou encore d'un assouplissement des règles d'urbanisme. Pour conclure, et en d'autres termes, monsieur le ministre, ne placez pas Notre-Dame « hors-la-loi » en

le présent projet de loi doit répondre à une situation exceptionnelle, sans se transformer en projet de loi d'exception. Il a vocation à permettre une réparation optimisée et diligente de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite de l'incendie du 15 avril dernier. pour ma part favorablement l'idée émise par ce texte de créer un établissement public, qui associera l'ensemble des partenaires : Ville de Paris, culte affectataire, mais aussi organismes collecteurs des dons, singulièrement le Centre des monuments nationaux, en charge de longue date de l'accueil payant du public dans les tours et parties hautes de la Il me semble également pertinent que les trois fondations privées siègent dans ce conseil d'administration, car elles seules peuvent représenter les donateurs. Je proposerai un amendement en ce sens. Je souhaite souligner qu'accepter la création d'un tel établissement public dédié ne préjuge pas de l'application des règles relatives aux procédures traditionnelles en matière de travaux sur monuments historiques. Bien entendu, nous exprimons notre refus de déroger aux règles légales et réglementaires des codes de l'urbanisme, de l'environnement, du patrimoine et des marchés publics. Si nous avons adopté ces règles dans notre droit positif, c'est qu'elles ont leur utilité ! Que diront demain d'autres maîtres d'ouvrage, publics ou privés, parisiens ou provinciaux, si l'on déroge ici, mais pas pour eux ? Cette disposition d'exception porte en elle le risque d'un détricotage de notre droit. C'est un danger inacceptable, non seulement pour notre patrimoine historique- les professionnels ont massivement exprimé ce sujet -, mais également pour notre urbanisme, nos paysages, notre protection écologique et la lutte contre tout favoritisme et toute corruption. Sur la question fiscale, je suis assez favorable à l'idée de passer de 66 % à 75 % de déductibilité jusqu'à 1 000 euros de dons. Ce geste n'impactera que très légèrement les recettes de l'État, dans la mesure où les recettes de TVA lors de la facturation des travaux seront pour leur part très importantes au regard des montants nécessaires à la restauration de l'édifice. Je terminerai mon propos en évoquant les fondations collectrices de dons, singulièrement la Fondation du patrimoine. Le remplacement de la collecte pour Notre-Dame de Paris par un appel aux dons Plus jamais ça ! » de nature généraliste au bénéfice d'une multitude de monuments en grave péril est destiné à protéger les missions traditionnelles de ladite fondation, puisque, des quatre organismes habilités à recueillir les dons de la souscription nationale, elle est la seule à bénéficier exclusivement de dons privés dans le champ unique de la protection du patrimoine. Les très nombreux correspondants bénévoles et délégués départementaux et régionaux de la fondation ont fait valoir le risque que leurs missions traditionnelles ne bénéficient plus des soutiens financiers nécessaires pour d'innombrables autres monuments qui souffrent dans la grande diversité de nos territoires, singulièrement ruraux- nous ne pouvons pas les oublier

dons a été à la fois surprenant et réconfortant et a révélé l'émotion et la solidarité des Français autour de ce monument inestimable.

l'éventuel différentiel, en plus ou en moins, qui pourrait à terme être constaté entre le montant des travaux et les sommes collectées. Des

l'égalité entre les personnes ayant fait des dons. Des règles comptables seront mises en place pour faire en sorte que les personnes ayant fait des dons le lundi 15 soient éligibles à la déduction

préciser que la souscription nationale est ouverte pour « le chantier » de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous nous direz,

autorise l'affectation d'une partie du produit de la souscription à la formation des professionnels. Il s'agit ici de tirer profit du drame de Notre-Dame pour mieux faire connaître les métiers du patrimoine qui connaissent actuellement une crise des vocations. Il ne faudrait pas que la référence au chantier qui est proposée par cet amendement

les fonds collectés par la souscription servent à la remise à niveau de l'enseignement professionnel, qui est une mission propre du ministère de l'éducation nationale.

À l'occasion de l'examen de l'article 2 qui précise la destination des fonds recueillis dans le cadre de la souscription nationale, je souhaiterais rappeler la situation préoccupante du secteur du patrimoine monumental depuis une quinzaine d'années : les crédits budgétaires qui lui sont destinés ont chuté de près de 40 %. Cette baisse drastique a conduit à l'arrêt de la restauration sur de nombreux chantiers, mais aussi à la fermeture de petites entreprises artisanales détentrices de savoir-faire pointus en matière de restauration, d'architecture et d'arts anciens. Ces savoir-faire sont parfois considérés comme perdus ; il est donc utile de prévoir la formation de professionnels afin de rénover des éléments datant de l'époque médiévale. L'article 2 dispose ainsi que les fonds collectés serviront au financement des travaux de restauration et de conservation de la cathédrale et à la formation de professionnels disposant des compétences requises. Je reste néanmoins dubitative quant à l'ajout, à l'Assemblée nationale, d'une référence à la formation «

qui précise notamment que ces travaux devront préserver l'intérêt historique, artistique et architectural de Notre-Dame conformément à la charte de Venise de 1964. disposons d'outils de formation de grande qualité. Le réseau des chambres des métiers et de l'artisanat a présenté au Gouvernement des propositions destinées à permettre aux artisans d'art d'accéder aux aux marchés de la restauration et à encourager la formation des jeunes. Chez les Compagnons du devoir, le système de formation est fondé sur l'apprentissage, mais aussi sur la transmission, valeur essentielle du compagnonnage, si bien que les savoir-faire se transmettent aussitôt

L'Assemblée nationale a inclus une disposition, selon laquelle les travaux doivent préserver « l'intérêt historique, artistique et architectural du monument ». C'est un premier pas apprécié.

la restauration de Notre-Dame ne doit pas concerner exclusivement le monument, mais aussi son intégration dans le paysage des rives de la Seine. Dois-je rappeler que la flèche de Notre-Dame a été pensée par Viollet-le-Duc et Lassus pour entrer en résonance visuelle avec la flèche de la Sainte-Chapelle,

le big data est une source d'informations éminemment précieuse pour la conduite de la restauration de la cathédrale. Preuve en est la mise en place d'une équipe de chercheurs dédiée du CNRS, qui va analyser très finement ces données. Cela va ainsi permettre une modélisation de la cathédrale en temps réel. Ce travail scientifique va évidemment intéresser les responsables du chantier de restauration, et, plus largement, les Parisiennes et les Parisiens, ainsi que tous les visiteurs français et Cette analyse des données va également permettre de faciliter demain la restauration d'autres lieux gothiques, dans des circonstances bien évidemment moins tragiques. Les simulations donneront aussi l'occasion de suivre l'évolution du chantier pas à pas.

en explorant la modélisation 3D de la cathédrale, suivant ainsi l'évolution du chantier. Évidemment, une visite virtuelle ne remplacera jamais la force du lieu, sublimement décrit par Charles Péguy, ou, plus près de nous, par Sylvain Tesson, mais cela permettra de ne pas couper l'édifice du reste du monde pendant ces quelques années. Le numérique est une passerelle, tant pour organiser une restauration pertinente de Notre-Dame de Paris que pour canaliser l'impatience légitime de ses très nombreux amis. La parole

part, je pense qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures : quand on donne une subvention, c'est toujours pour l'investissement et rarement pour le fonctionnement. En l'occurrence, je pense que l'entretien doit rester à la charge de l'État et non de la générosité privée.

Ensuite, comment réhabiliter ? Une fois n'est pas coutume, je partage le point de vue de notre collègue Assouline à cet égard. Le Sénat est là pour mettre des garde-fous.

En effet, je ne pense pas que les donateurs aient eu comme intention de financer les frais de fonctionnement de l'établissement public, même si, on l'a bien compris, celui-ci vise à coordonner la reconstruction de

Il s'agit de précisions qui me semblent fort utiles et de nature à rassurer les donateurs sur la manière dont seront utilisées les sommes qu'ils ont versées. Le produit de la souscription doit évidemment permettre de réparer les dommages causés par le sinistre du 15 avril, et non de financer des de financer des dépenses qui incombent à l'État, en tant que propriétaire du monument. Je doute d'ailleurs que les donateurs aient jamais eu à l'esprit que leurs dons puissent servir à financer les salaires, loyers ou dépenses d'entretien et de fournitures d'un nouvel établissement public, quand bien même serait-il chargé de la maîtrise d'ouvrage de Notre-Dame.

Monsieur Retailleau, vous avez une connaissance très fine de la volonté de chaque donateur de Notre-Dame de Paris. Bravo ! Vous avez dû les consulter les uns après les autres pour savoir exactement quelle était leur volonté individuelle

en partie, avec l'article 2 : « Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier, dont l'État est propriétaire, ainsi qu'à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui sont requises pour ces

Il faut savoir qu'entre le relevé intégral de la charpente réalisé par Viollet-le-Duc et aujourd'hui, très peu d'observations archéologiques ont été réalisées sur cette charpente.

que l'investissement programmatique de recherche sur ce monument soit exceptionnel. Sur ce point, nous aimerions avoir des engagements de votre part. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

nous voulons réaffirmer que le ministère de la culture ne saurait s'exonérer de ses missions traditionnelles, qu'il doit assumer.

d'échafaudages sur la cathédrale ou le retrait définitif des statues d'apôtres qui ornaient la base de la flèche et qui avaient été déposées quelques jours avant le sinistre. J'exagère peut-être un peu ... Par ailleurs, et surtout, cette formulation laisse entendre que la cathédrale ne peut subir un iota de modification ne peut être restaurée avec une once d'imagination. Nous n'aurions jamais eu la flèche de Viollet-le-Duc si une telle disposition avait été prévue dans un cahier des charges antérieur au démontage, pendant la Révolution, de la première flèche de 1250. Si une telle disposition s'était appliquée au Louvre, François Mitterrand n'aurait jamais pu faire aménager le Grand Louvre et son entrée par la pyramide de l'architecte Ming Pei, tout récemment disparu.

Nous ne pouvons pas ignorer que la présence de la cathédrale Notre-Dame a été déterminante dans le classement du site « Paris, rives de la Seine », comme l'a rappelé Mme la présidente de la commission. Or la France, en ratifiant la convention du patrimoine mondial, s'est engagée à respecter un certain nombre de principes.

et pourrait nous contraindre à certains travaux, je pense notamment à la nature des voûtes et des murs. comme l'usage des matériaux dépend de leur disponibilité, il me semble préférable de nous en tenir à la nécessité de préserver le monument dans son dernier état visuel-

car il me paraît de nature à éclairer les choix retenus pour la restauration de Notre-Dame. Il permettra de comprendre les raisons techniques ou sécuritaires qui justifient,

cette espèce de défiance, de méfiance permanente vis-à-vis de l'État et de ses serviteurs ? Franchement, le chef de l'État

relire une phrase : « Les couches d'histoire acquises au fil du temps par un bien culturel sont considérées comme des attributs authentiques de ce bien culturel. » Cela veut dire que la flèche de Viollet-le-Duc est constitutive de ce monument dont l'histoire va

le principe de la charte de Venise, de revenir au bâtiment tel qu'il était avant d'être détruit par l'incendie. Bien évidemment, le Parlement ne doit pas dire ce qu'est le beau et le vrai. Les essais d'art officiel n'ont jamais été très concluants ! Ce qui est essentiel, c'est que le Parlement fasse respecter des principes d'éthique que nous défendons avec force à l'échelle internationale. La discussion sur la flèche de Viollet-le-Duc doit entrer dans ce débat éthique sur des valeurs que nous portons dans le monde. Je voterai moi aussi les amendements de notre collègue Leleux, parce qu'ils sont conformes aux engagements internationaux de la France.

mérite de dépasser ces querelles politiciennes pour faire consensus. Et je regrette, monsieur le ministre, que ce projet de loi ne fasse pas consensus entre vous et nous et, qui plus est, avec l'Assemblée nationale. Si nous avons déposé cet

Monsieur le ministre, je ne vais pas employer les mêmes termes que mon collègue, mais je vous trouve bien sévère envers le Sénat. Tout le monde a dit à peu près la même chose, c'est-à-dire que cela relève du travail parlementaire. Je vous renvoie au début de cet article. Personne

Pierre Rosenberg, que personne ne contestera ici, avait l'habitude de dire que le XIX siècle était « le » grand siècle, notamment pour la sculpture et la peinture. Regardez ce que le XIX siècle nous a apporté en peinture

Viollet-le-Duc est un grand architecte. On cite souvent Hugo comme quelqu'un qui a contribué à sauver Notre-Dame. Je pense que Viollet-le-Duc a tout autant contribué contribué à sauver la cathédrale que Hugo. Je pense qu'aucune indignité artistique et culturelle ne doit peser ni sur le XIX siècle- qui est un siècle récent

Je suis tout simplement un admirateur quasi inconditionnel de l'oeuvre de Viollet-le-Duc et de Lassus. Pardonnez-moi, je crains simplement que le fait de remplacer cette architecture admirable puisse dénaturer au fond l'ensemble

Le scrutin est ouvert.

Cidrac. Cet amendement prévoit un décret, dont le but sera d'éclaircir les conditions de formation des professionnels pouvant concourir à la restauration et à la conservation de Notre-Dame. L'article 2 mentionne bien des compétences particulières, mais il ne les précise pas.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 3 prévoit que, au-delà du Trésor public, quatre opérateurs sont chargés de recueillir les fonds destinés à la conservation et à la restauration de Notre-Dame.

entre ces organismes collecteurs et le maître d'ouvrage délégué. En outre, les versements ne se feront que sur appel de fonds au fur et à mesure de l'avancée du chantier et des besoins en travaux. Ces conventions seront garantes des intentions des donateurs.

votre étude d'impact, on a le sentiment que la création du nouvel établissement se justifie uniquement par la volonté d'assurer une gouvernance spécifique.

Il va falloir recevoir ces visiteurs dans les meilleures conditions de sécurité et d'accueil. De plus, il faudra sans doute organiser des offices. Il serait également opportun d'organiser des expositions sur l'état d'avancement du chantier, voire de présenter les collections d'art- trésors, tableaux et statues -qui ont échappé au sinistre. il semble utile et sage de prévoir dès à présent un aménagement des abords du parvis, qui, en toute logique, doit lui aussi être financé par la générosité nationale. Ce projet s'inscrit dans la continuité de la restauration de Notre-Dame.

très sensible à la plaidoirie de notre collègue David Assouline. Il a raison : le parvis de la cathédrale ne peut pas être considéré comme extérieur à ce qui s'est passé et il faudra intervenir

que la question des abords et singulièrement du parvis, de son animation, de l'appropriation progressive des travaux de restauration du monument par la population parisienne et au-delà, ne peut